rapport. Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute. Monsieur le ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur de la mission d'information qui a demandé ce débat. Madame la présidente,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine ont mis en relief les fragilités de notre économie. Ainsi, l'incapacité de la France, patrie de Pasteur, à développer un vaccin contre le covid-19 nous a brutalement rappelé que nous ne faisions plus partie des États leaders dans l'innovation. Sommes-nous pour autant condamnés à jouer le rôle de fournisseur d'innovations technologiques de qualité et bon marché, transformées par des entreprises étrangères en innovations industrielles, nous revenant sous forme d'importations néfastes à notre balance commerciale ? Ce n'est pas ce que nous souhaitons. La crise énergétique pourrait évidemment aggraver le phénomène, puisqu'elle rend plus difficile la réimpatriation des chaînes de production.

en effet que nous comprenons tous, chacun avec sa sensibilité politique, le drame industriel qui s'est joué dans notre pays. J'en profite pour remercier chaleureusement tous les membres de la mission qui m'ont accompagnée au cours de ce travail et qui l'ont enrichi de leur expérience propre et des exemples issus de leur territoire, singulièrement son président Christian Redon-Sarrazy, qui a su nous faire profiter de sa connaissance de ces sujets, notamment pour ce qui concerne la formation dans les territoires. Nous avons tout d'abord constaté un paradoxe- en France, on adore les paradoxes ! -, à savoir que notre pays investissait massivement en faveur de l'innovation pour des performances industrielles qui n'étaient pas vraiment à la hauteur. Pourtant, il n'y a pas de : la France dispose des atouts nécessaires pour être une économie de rupture technologique, créatrice d'emplois dans les territoires. Il s'agit de tenir compte des « erreurs françaises » qui ont jusqu'à présent empêché de transformer mieux l'essai de l'innovation industrielle, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour que la France redevienne une nation industrielle innovante et souveraine. Deux principes ont guidé l'élaboration de nos recommandations : l'efficacité de la dépense publique et le caractère opérationnel des mesures proposées. Le soutien de la croissance et du développement des industries innovantes est l'affaire de tous, et seule une action coordonnée du Parlement, du Gouvernement et des acteurs privés permettra de relever les défis auxquels notre pays doit faire Le Parlement a un rôle essentiel à jouer. Deux tiers des dépenses de soutien à l'innovation sont des incitations fiscales, notamment avec le crédit d'impôt recherche (CIR) qui représente une dépense annuelle de 6,6 milliards d'euros. son efficacité est inversement proportionnelle à la taille des entreprises bénéficiaires : véritable incitation à l'innovation pour les petites et moyennes entreprises (PME), il est trop souvent, pour certains grands groupes, une forme d'aubaine fiscale.

nous souhaitons supprimer le taux de 5 % de CIR au-delà du plafond de 100 millions d'euros de dépenses de R&D, tout en augmentant à due concurrence le taux en deçà de ce plafond.

Dire que, sans cette mesure, nos grands groupes délocaliseront leurs activités de recherche ou que nous n'attirerons plus les investisseurs étrangers est un chantage à l'emploi

Nombre d'entreprises consolident leurs résultats pour déterminer leur bénéfice global en compensant les pertes de certaines filiales avec les résultats positifs des autres afin de diminuer leur impôt sur les sociétés. Or, même dans cette hypothèse, le CIR peut être calculé au niveau de chaque filiale. filiale. L'équité fiscale exige qu'en cas d'intégration fiscale le crédit d'impôt soit également calculé au niveau de la holding, et non dans chaque filiale. Selon les calculs du Comité Richelieu, une telle réforme

que, depuis que nous avons publié nos recommandations, ce sont bien les ajustements à la marge que nous proposons, au nom de l'efficacité de la dépense publique, qui focalisent l'attention, alors même que nous approuvons la sanctuarisation du CIR. C'est pourquoi C'est pourquoi il m'a paru important de concentrer mon propos sur ce sujet afin de lever tout malentendu. Le président de la mission d'information aura tout loisir, en conclusion de ce débat, de revenir sur les autres mesures, nombreuses, que nous Je tiens à évoquer, dans le temps qui me reste, quelques pistes d'action qui ne relèvent pas du Parlement, mais qui sont à la main du Gouvernement. Un principe, d'abord : préférer le chiffre d'affaires aux subventions, en mobilisant la commande publique au service des entreprises industrielles innovantes. Une règle d'or, ensuite : faciliter les démarches administratives raccourcir les délais. C'est avant tout une question de volonté politique. L'exemple du terminal méthanier flottant au Havre, dont la construction devrait commencer six mois à peine après que ce projet a été envisagé, montre que nous pouvons le faire

pointe les lacunes de notre industrie et présente des pistes pour permettre à la France de redevenir une nation industrielle, innovante et souveraine. Notre pays subit en quelque sorte les conséquences de la croyance, à l'oeuvre dans les années selon laquelle il était possible de décloisonner les activités de production de celles de conception et d'innovation, et de créer en quelque sorte une entreprise sans usine. Suivant cette croyance, l'industrie française a ainsi délocalisé une grande partie de ses moyens de production, détruisant dans le même temps des millions d'emplois industriels sur plusieurs décennies- près de 3 millions d'emplois entre 1975 et 2014. L'inefficacité de ce décloisonnement est aussi mise en exergue par la faible corrélation, révélée par le rapport d'information, entre le soutien public massif à l'innovation à l'innovation et l'incapacité de la France à faire émerger, dans le même temps, de nouveaux champions industriels. Sans l'industrie, nous ne serons pas en mesure de redevenir une grande nation d'innovation. Industrialisation et innovation sont deux combats qu'il nous faut mener de front, de manière simultanée. C'est une nécessité comprise au plus haut sommet de l'État, puisque différents plans ont été déployés à l'échelon national depuis 2017 afin d'engager la reconquête industrielle de la France. des crises extérieures nous ont bousculés. La crise sanitaire a révélé notre extrême dépendance et a mis en lumière les faiblesses de notre modèle industriel, notamment sa dépendance aux importations. la même façon, avec la crise ukrainienne, l'Union européenne a pris conscience qu'elle avait besoin de réduire sa dépendance énergétique, de conserver la maîtrise de ses décisions et de construire la « souveraineté européenne ». Enfin, l'urgence climatique est là. L'été 2022 a vu se multiplier les catastrophes liées au réchauffement climatique. Il faut mettre notre dépendance aux énergies fossiles derrière nous. Pour atteindre 40 % d'électricité issue d'énergies renouvelables à l'horizon 2030, nous devons diversifier notre mix énergétique. Biométhane, biomasse, hydrogène décarboné, éolien en mer, photovoltaïsme, exploitation de l'énergie des courants des marées : un énorme potentiel technologique et industriel s'offre à nous. La crise sanitaire, le conflit ukrainien et l'urgence climatique agissent comme des accélérateurs accélérateurs d'innovations. Ces défis nous poussent à faire preuve de courage, d'audace et d'inventivité. Nous devons nous donner l'ambition de construire nos rêves. C'est l'objectif de France 2030 : une ambition publique pour répondre aux défis écologique, démographique, économique, industriel et social d'un monde en perpétuelle évolution. Ce sont ainsi 34 milliards d'euros qui ont été investis pour qu'en France les entreprises, les universités et les organismes de recherche réussissent pleinement leur transition vers les filières stratégiques. En amont, nous devons mettre les bouchées doubles sur la formation et l'apprentissage, les nouvelles filières, nos écoles et nos organismes de recherche dans des segments de pointe. En cours de processus, il faut permettre à une start-up qui débute ses recherches de monter rapidement ses prototypes. Au bout de la chaîne, c'est la réindustrialisation de nos territoires elle a commencé, elle doit être renforcée. Je ne citerai qu'un exemple, celui de STMicroelectronics à Crolles. C'est, à mon sens, le symbole que la réindustrialisation est possible quand la volonté politique est là. Ce ne sont en effet pas moins de 6 milliards d'euros qui ont été investis sur ce site, où la France va installer la plus grande unité de production de semi-conducteurs en Europe et créer plus de 1 000 emplois supplémentaires. Cet exemple est le symbole de la France du savoir et de la recherche, ainsi que de notre reconquête industrielle. Le groupe RDPI se tiendra au côté du Gouvernement et de tous ceux

mes chers collègues, je tiens à mon tour à saluer le travail de qualité mené par la mission d'information, dont la technicité et la précision n'ont jamais fait défaut.

Le système français doit considérablement améliorer l'innovation et en faire l'une de ses priorités. Les propositions de la mission d'information vont dans ce sens et gagnent à être entendues par les pouvoirs publics. Le problème ne se limite toutefois pas à la France. La dimension européenne ne doit pas être oubliée. L'Union européenne doit même reprendre le leadership sur l'innovation de rupture. Face aux avances technologiques prises ou en passe de l'être par des puissances émergentes telles que la Chine, comment faire de l'Union européenne une puissance qui résiste ? Prenons l'exemple de la 5G. La législation française est adaptée au contexte, mais il convient de rester attentif à l'évolution des risques sur l'ensemble du territoire européen. Tous les pays n'ont pas le même niveau d'expertise sur ces questions. Il convient donc non seulement de soutenir la mise en oeuvre de la boîte à outils de l'Union européenne susceptible de faciliter l'application de mesures nationales dans le domaine de la 5G et de veiller à l'évolution des risques, de soutenir la réalisation du projet Hexa-X et d'autres initiatives et financements communautaires susceptibles de favoriser l'émergence d'acteurs européens de premier plan dans le domaine de la 6G. Soutenir, mais comment ?

La capacité de la France et de l'Union européenne à soutenir l'émergence d'acteurs européens alternatifs est certainement l'une des conditions pour garantir notre souveraineté. domaine spatial, l'Union européenne doit se donner les moyens de rester un acteur majeur. Front de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, l'espace est l'un des enjeux de la course pour la place de première puissance mondiale entre Washington et Pékin. La Chine est devenue une puissance spatiale majeure, qui mène de front des programmes d'exploration lunaire et martienne, des vols habités, des lancements de satellites à vocation scientifique, commerciale ou militaire, et même la construction d'une station spatiale chinoise.

définir une politique nationale et une politique communautaire qui prennent en compte les récents développements des ambitions chinoises.

Plus largement, il faut réaffirmer la nécessité d'une recherche publique forte, laquelle ne peut s'accommoder d'un enseignement supérieur en berne, comme c'est le cas aujourd'hui et depuis si longtemps. l'Union européenne doit encourager le développement d'un secteur privé performant en mettant en place les conditions optimales à la croissance des start-up innovantes. C'est l'application cumulative de ces quatre grands axes qui permettra de favoriser l'innovation et la compétitivité. Le rapport de la mission d'information va dans ce sens. La plupart de ses préconisations sont une déclinaison de ces quatre axes. Faire de la commande publique un levier essentiel de croissance pour les entreprises industrielles innovantes ? C'est le deuxième axe. Faire de la propriété industrielle et de la normalisation des sources de compétitivité ? C'est le premier axe. Inciter les grands groupes à s'impliquer dans l'émergence et la croissance des entreprises innovantes ? C'est le Élaborer dès 2022 une loi pluriannuelle de programmation de l'innovation pour renforcer l'efficacité de la politique de valorisation ? C'est le J'en viens à un point extrêmement important, qui a été mis en exergue. Nous préconisons de systématiser les évaluations des politiques de transfert et de valorisation menées par les organismes publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et de confier cette nouvelle mission au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Oui, l'évaluation doit être une priorité majeure de nos politiques publiques. Elle est en même temps un enjeu essentiel et une culture que nous ne possédons pas, ce qui est bien dommage. Sans évaluation, l'attribution des financements sera naturellement fléchée vers les acteurs déjà installés, favorisant les consortiums qui bénéficient déjà d'un soutien européen. Ces derniers ne sont

On sécurise pour que le résultat en 2025 soit ce que l'on voulait en 2022, mais le monde aura changé trois fois entre-temps et on risque de tomber à côté. d'information indique que nous devons réorienter les aides fiscales pour mieux accompagner le passage à l'échelle des petites et moyennes entreprises innovantes,

d'évasion et d'optimisation fiscales, si souvent dénoncées, et pour endiguer son détournement par des bénéficiaires insuffisamment contrôlés. Enfin, pour aller jusqu'au bout de l'évaluation, interrogeons-nous sur le rôle que nous devons donner au Parlement dans les transformations que nous préconisons de mettre en oeuvre. N'oublions pas le Parlement, car il a toute sa place ! Sur le modèle de la Darpa (), l'agence du département de la défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies qui rend des comptes au Sénat américain,

Merci à nos collègues qui ont entrepris cette démarche, nous permettant ainsi de débattre et, je l'espère, d'oeuvrer à un sursaut bien nécessaire de la politique d'innovation de notre pays.

d'information complète celui qui a été examiné hier soir sur la souveraineté économique et l'indispensable réindustrialisation. Oui, relancer l'innovation est essentiel pour la souveraineté de la France et pour la capacité de notre pays à maîtriser son destin et son avenir.

Force est de constater que d'énormes retards ont été accumulés et qu'inverser les tendances négatives qui ont prévalu depuis près de trente ans exige un véritable sursaut collectif, une mobilisation générale et des interventions publiques

Ce terreau, c'est une appétence pour la science, ainsi qu'un haut niveau scientifique et technique de nos concitoyens et de notre jeunesse. Comment ne pas être alarmé par la rapide détérioration

L'affaire n'est pas nouvelle : le rapport Villani-Torossian le disait déjà, mais les dispositions prises en 2018 n'ont pas suffi à redresser la barre.

Plus largement, la situation de l'enseignement supérieur est elle aussi alarmante. J'approuve la demande d'une loi de programmation pluriannuelle, à condition- mais je sais que telle n'est pas l'intention du président et de la rapporteure

dans notre hémicycle, nous étions nombreux à estimer que les montants étaient insuffisants et qu'ils ne permettraient pas d'atteindre 3 % de PIB pour la recherche et 1 % pour la recherche publique. Nous sommes actuellement tout juste dans la moyenne européenne, bien loin derrière l'Allemagne. C'est pourtant un point majeur pour la compétitivité de la France, sans doute bien plus important que l'obsédante

pas. La trajectoire d'emplois est nettement inférieure, puisque seuls 376 emplois ont été créés contre les 700 prévus. Sans chercheurs, comment innover ?

en effet de l'innovation que découlent les nouvelles sources de croissance de notre économie, la bonne santé de nos entreprises, la vitalité de nos territoires et le progrès humain. Face au caractère inéluctable du changement climatique, il nous est imposé de changer nos modes de production afin de restreindre leurs effets néfastes sur l'environnement et d'atteindre les objectifs bas-carbone à horizon 2050. Dans une politique visionnaire, nos prédécesseurs nous ont légué le fruit inestimable d'une innovation tout à fait remarquable, une production électrique quasiment décarbonée, nous plaçant de fait parmi les nations les plus avancées du monde en la matière. La crise sanitaire a agi comme un puissant révélateur de notre manque de capacités d'innovation. Notre pays a connu une saignée industrielle extrêmement douloureuse à partir des années 1980, dont nous payons toujours les conséquences en termes d'emploi, de cohésion territoriale et de prospérité. La nécessaire réindustrialisation de notre pays et l'adaptation au climat ne peuvent passer que par un effort puissant en faveur de la recherche et de l'innovation. Depuis le début des années 2000, la France a su accroître le volume du soutien public à l'innovation, qui est passé de 3,5 à 8,7 milliards d'euros par an en quinze ans. Au total, 110 milliards d'euros seront mobilisés

La France compte désormais 20 000 start-up et 27 licornes. Une seule est une start-up industrielle. L'innovation bénéficie donc en majeure partie au secteur du numérique. La mission d'information à laquelle j'ai eu la chance de participer propose plusieurs voies d'action, qui, je le crois, permettront à l'innovation et à la recherche de redevenir le centre de gravité de notre économie. notre vision est trop linéaire. Elle conduit les pouvoirs publics à soutenir l'innovation essentiellement au travers d'appels à projets qui ne permettent ni de construire des feuilles de route industrielle et technologique ni d'avoir une vision de long terme. Avant toute mesure paramétrique et sectorielle, il convient de résoudre la problématique que représente l'enseignement scientifique dans notre pays. Les besoins de l'économie française en termes de nouveaux ingénieurs sont estimés entre 50 000 et 60 000 chaque année ; or nos écoles n'en forment que 33 000 par an. Ce différentiel contribue à un affaissement de notre compétitivité. Pour rester une grande puissance innovante et industrielle, il faut dès maintenant s'attaquer à la question de l'enseignement des sciences dans notre pays. Si l'on en croit les statistiques du ministère de l'éducation nationale, « le niveau des élèves de 4 en 2019 en maths est équivalent à celui des élèves de 5 en 1995 Il nous faut inverser la tendance. Une hausse des rémunérations des enseignants et des chercheurs ainsi qu'une loi de programmation de l'enseignement supérieur sont indispensables pour relever le niveau de l'enseignement, susciter des vocations d'ingénieurs, de doctorants, de scientifiques, attirer et conserver nos talents. Le lien entre innovation et industrie est fondamental. Ainsi, 70 % de la recherche privée en France est réalisée par l'industrie manufacturière. Il est donc essentiel d'orienter l'innovation vers la réindustrialisation en favorisant les partenariats entre centres de recherche publics et privés et en permettant à un nombre accru d'entreprises, notamment les petites, de se saisir des dispositifs de soutien existants. Il convient également d'organiser des transferts de technologie vers des entreprises françaises produisant sur le sol national. Dans cet esprit d'encouragement de l'innovation, il est impossible de ne pas évoquer le crédit d'impôt recherche. Je serai cependant bref sur le sujet, car vous l'avez longuement

d'un recalibrage du CIR vers les bénéficiaires en ayant le plus besoin. La mission d'information propose de doubler le plafond du crédit d'impôt innovation pour le porter à 800 000 euros

que nous nous sommes imposées, année après année, rendant la vie de nos entreprises de plus en plus difficile. Il est anormal qu'un laboratoire de thérapie génique, secteur innovant par excellence, puisse

c'est tout le pays qu'il nous faut remettre en état de marche, à commencer par notre jeunesse, pour lui donner le goût de la découverte et de l'expérimentation scientifique. Il nous faut accompagner les entreprises innovantes financièrement, mais aussi engager la puissance publique dans un rôle de facilitation de l'innovation. Les leviers à activer sont nombreux : utiliser la commande publique pour favoriser l'innovation, simplifier les procédures administratives, affiner les dispositifs fiscaux existants et faciliter le financement privé de l'innovation.

dans le cadre de la mission d'information « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l'erreur française ». Lorsque le groupe Les Indépendants - République et Territoires a pris l'initiative de créer une mission d'information sur ce thème, nous avons été curieux et enthousiastes à l'idée de débusquer des réponses à ce qui pouvait s'apparenter à un paradoxe à la française. Force est de constater que des faits historiques, culturels, politiques, économiques et financiers sont venus enrichir nos interrogations initiales-

Par conséquent, il conviendrait de renoncer à cette conception mercantile de l'enseignement supérieur et de la recherche et de considérer qu'il s'agit d'un investissement pour l'avenir, afin de former celles et ceux qui intégreront les exécutifs de potentielles futures industries.

En somme, toutes les recommandations formulées dans le rapport d'information revêtent une grande importance, mais certaines nous paraissent particulièrement saillantes. Je pense d'abord à l'augmentation du nombre de « sites industriels clés en main » par une meilleure planification de leur utilisation.

l'adoption de critères économiques, écologiques, sociaux et de souveraineté pour évaluer l'objectif de promotion du transfert technologique et de l'innovation, qui est fondamentale. Il s'agit de permettre à ce secteur de relever les défis qui s'imposent à la société tout entière.

Je me réjouis que soient évoqués à plusieurs reprises tout au long du rapport d'information la situation et le rôle singulier des PME et des ETI face à l'innovation. quatre points qui ont particulièrement retenu mon attention. Premièrement, il faut renforcer la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'innovation et l'entrepreneuriat devraient être encouragés dès l'école, les formations à l'entrepreneuriat généralisées dans l'enseignement supérieur. Il faut mettre fin à la culture de la peur de l'échec, de la honte, afin d'encourager la créativité et l'innovation. Relancer l'esprit d'entreprise est crucial, dans un pays qui glisse sur la pente dangereuse de l'assistanat. Deuxièmement, il faut faire converger le temps administratif et le temps économique. Il faut intégrer le temps de l'entreprise dans les procédures administratives, mettre en place des procédures rapides pour agir et adopter des lois pluriannuelles pour sécuriser l'environnement juridique des entreprises.

Les PME pourraient ainsi enfin accéder à la commande publique, qui représente des montants considérables. Le triplement du plafond de l'achat innovant irait également dans le bon sens. Plus généralement, ce qui ressort du rapport d'information, c'est la nécessaire simplification des procédures administratives. Les entreprises ont besoin de pragmatisme, de lisibilité, de simplicité ! En 2010, selon l'OCDE, les charges administratives représentaient 3 % du PIB de la France, soit 60 milliards d'euros. Aujourd'hui,

et une recommandations. Une simplification ambitieuse des démarches des entreprises favoriserait la création et la croissance des entreprises, et par là même l'innovation réorienter les aides fiscales et financières. On ne peut en effet penser innovation sans mettre en place un environnement fiscal, financier et économique adapté.

Si la fiscalité et le soutien public ont évidemment leur rôle à jouer, l'investissement privé doit en être le complément. La posture de nos grandes entreprises vis-à-vis de nos start-up et PME doit évoluer. Les grands groupes n'aident pas nos petites entreprises. L'inscription de ce critère dans la RSE serait une excellente chose, afin que ces grands groupes soient plus que des « grands frères bienveillants ». Monsieur le ministre, j'insisterai enfin sur le caractère interministériel du sujet. On ne peut penser innovation et recherche sans intégrer le développement économique. Sans débouchés pour nos chercheurs, pour nos innovations, le risque, comme on l'a malheureusement déjà constaté, c'est la fuite de nos cerveaux et le déclassement de nos entreprises en raison de l'obsolescence technologique.

le financement de la recherche publique et de la recherche privée stagne autour de 2,2 % du produit intérieur brut, à tel point que nous avons abandonné à d'autres pays européens le leadership en matière de R&D.

l'objectif étant de parvenir à un effort national de recherche équivalent à 3 % du PIB. Cette loi prévoyait également de renforcer l'attractivité des métiers scientifiques, de consolider les dispositifs d'évaluation, d'organisation et de financement de la recherche et de faciliter la diffusion de la recherche dans l'économie et la société. Lors de l'examen de ce texte, j'avais affiché un optimisme très relatif tant la trajectoire budgétaire me semblait peu crédible et surtout peu efficace au regard de l'importance de l'écart de compétitivité à combler entre notre pays et les pays européens les plus avancés en matière de recherche et d'innovation. C'est d'ailleurs sur l'initiative du Sénat que l'intensité de l'effort budgétaire a été renforcée sur les premières années de la programmation. J'avais en outre émis des doutes sur la capacité de cette loi à fixer un cadre réellement motivant pour nos chercheurs et enseignants-chercheurs, susceptible de favoriser leurs activités de recherche en France et non à l'étranger. L'absence de vision sur ce que doit être la politique publique de recherche à moyen et long termes y est sans doute pour beaucoup ... La commission de la culture du Sénat a récemment rendu public son rapport d'information sur la mise en oeuvre de la LPR. Le bilan que nous avons dressé démontre que ce texte était nécessaire, mais que son application sur le terrain reste perfectible. a permis un bon début de réinvestissement public dans la recherche, sa durée- dix ans -et l'intensité de l'effort budgétaire doivent néanmoins être reconsidérées, d'autant que cet effort est aujourd'hui très largement absorbé par l'inflation.

-juge pour sa part nécessaire de considérer la recherche comme un investissement de long terme dans l'innovation. Trop longtemps, hélas, l'investissement public dans la recherche a été perçu comme un coût et celle-ci a, de ce fait, régulièrement fait fonction de variable d'ajustement pour réduire le déficit budgétaire de l'État.

Par ailleurs, la politique de rémunération des chercheurs doit être plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui si nous voulons retenir nos meilleurs chercheurs et attirer les talents étrangers à fort potentiel. Le cas d'Emmanuelle Charpentier, jeune prix Nobel de chimie, partie mener ses recherches pionnières et majeures hors de France, n'est pas anecdotique : quand un chercheur de ce niveau fait le choix de poursuivre ses recherches à l'étranger, il emporte avec lui son aura, ses financements ses compétences. En outre, il ne fera pas bénéficier de jeunes chercheurs français de l'étendue de ses connaissances. Je suis pour ma part assez optimiste pour l'avenir, même s'il nous faudra persister dans notre effort budgétaire. En effet, le réinvestissement dans la recherche est en marche.

Les budgets en croissance offrent de nouvelles perspectives d'accompagnement des communautés scientifiques. Les premiers résultats sont là : le taux de succès aux appels à projets génériques atteint désormais plus de 23 % et le taux de préciput est passé de 19 % en 2020 à 25 % en 2021. En outre, le soutien à la recherche partenariale a été considérablement renforcé. Nous savons qu'il s'agit d'un puissant levier en faveur de l'innovation. En conclusion, j'évoquerai trois enjeux majeurs auxquels nous devrons apporter une réponse singulière et courageuse. Il nous faudra tout d'abord procéder à une clarification du paysage français de la recherche. Celui-ci est en effet constitué d'une pluralité d'acteurs- organismes nationaux de recherche, établissements d'enseignement supérieur, agences de financement, unités mixtes de recherche -, dont les missions ne sont pas forcément bien réparties et les relations pas toujours fluides. Il nous faudra ensuite donner un cap à la recherche française. La programmation budgétaire de la LPR n'a pas été accompagnée d'une programmation stratégique et c'est incontestablement l'une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a modérément adhéré à la réforme promue par le Gouvernement. Il nous faudra enfin favoriser une meilleure articulation entre recherche publique et secteur privé, et ce dès l'amorce des projets de recherche, car il n'y a pas d'innovation sans recherche fondamentale. Si nous sommes capables de répondre à ces trois enjeux, la France redeviendra un grand pays innovant dans tous les secteurs d'avenir- systèmes numérisés, nanotechnologies, nouvelles énergies, biologie, santé

Voilà plusieurs décennies que la France s'est engagée sur la voie de la désindustrialisation. Nous avons laissé partir nos usines, ne gardant ici que les centres de décision. C'était le rêve de la mondialisation heureuse ! Résultat : nous n'avons plus guère d'usines, nous exportons nos cerveaux et nous importons les produits que ces mêmes cerveaux, formés sur deniers publics, fabriquent à l'étranger. Nous sommes perdants sur toute la chaîne de valeur. Ce qui est heureux toutefois, c'est que nous en sommes désormais conscients. Il aura fallu plusieurs crises, singulièrement la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, pour nous en rendre compte : nous avons perdu notre souveraineté industrielle. L'objectif fait maintenant consensus : il faut réindustrialiser le pays. C'est bon pour nos importations, bon pour nos emplois, bon pour la transition énergétique, bon pour la cohésion sociale. La bataille théorique a été gagnée. Nous devons désormais passer à la pratique. Or, en la matière, les choses se compliquent : d'abord parce qu'il faut analyser précisément les causes de notre déclin industriel, ensuite, parce qu'il faut identifier des remèdes pour guérir le mal-et c'est souvent là que le bât blesse. C'est pourquoi je me réjouis que le groupe Les Indépendants - République et Territoires, auquel j'appartiens, ait créé cette mission d'information, qui visait précisément à identifier les principaux blocages empêchant notre pays de convertir ses innovations scientifiques en innovations industrielles. Je tiens à saluer l'engagement de Vanina Paoli-Gagin, qui est à l'origine de cette initiative et qui a accompli un travail de fond pour auditionner de très nombreux acteurs et proposer des solutions opérationnelles et concrètes pour relever cet immense défi. Ce travail a porté ses fruits : toutes les recommandations ont été adoptées à l'unanimité. C'est dire s'il y a consensus sur le sujet. Je ne reviendrai pas en détail sur chacune d'elles. Le rapporteur a déjà rappelé les principales mesures, notamment fiscales, pour transformer l'essai de l'innovation. Je me contenterai de tirer deux leçons du rapport d'information. La première leçon concerne la relation entre science et entreprise. Transformer l'essai de l'innovation, c'est traduire les avancées scientifiques en solutions opérationnelles, c'est faire le lien entre la recherche fondamentale et les projets industriels, entre le monde académique et le monde de l'entreprise. À cet égard, notre université recèle encore de très puissants éléments de conservatisme. Il n'est pas rare d'y croiser des enseignants et des chercheurs qui soutiennent mordicus que la recherche, pour rester pure, ne doit surtout pas trouver d'application concrète, que tout transfert de propriété intellectuelle ou tout brevet déposé avec une entreprise est une compromission terrible avec le Grand Capital. Ces réflexes corporatistes découragent encore trop souvent les vocations de ceux qui veulent valoriser autrement leurs savoirs. Et pour cause : une incursion dans le monde de l'entreprise est parfois perçue par les chercheurs comme un égarement de carrière, qui peut pénaliser l'avancement au sein de l'université. Il faut donc repenser le modèle académique pour permettre de mieux appréhender ces trajectoires, qui sont enrichissantes, à la fois pour nos chercheurs et pour nos universités.

La seconde leçon que je tire du rapport d'information, c'est l'absolue nécessité de simplifier notre bureaucratie. Nos entrepreneurs, mais aussi nos universités, nos chercheurs, nos laboratoires, tout l'écosystème l'affirme sans ambages : la France est un Absurdistan, où le formulaire est la norme et l'administration l'arbitre de tout. Nous avons laissé se développer tout un ensemble de règles qui nous étouffent. Le rapport d'information l'illustre par un exemple éloquent : pour démarrer l'activité d'un laboratoire de thérapie génique, il faut attendre près de dix mois en France. En Suisse, on part du principe que tout est en règle et l'entreprise peut commencer à produire cependant que le dossier est instruit en bonne et due forme. Voilà ce que nous devons faire en France : miser sur la confiance et remettre l'administration au service des usagers. C'est non pas aux Français, notamment aux entrepreneurs, qui prennent des risques pour faire bouger les choses, de s'adapter à l'administration, mais bien à l'administration de s'adapter à eux. Il est aberrant de financer par nos impôts des délais qui font perdre de l'argent à la collectivité. Pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place des instruments très efficaces, notamment parce qu'ils étaient immédiatement opérationnels. Bien sûr, il y a eu des erreurs et parfois des abus, mais y en a-t-il plus lorsque la défiance prévaut au sein de l'administration ? À mon avis, non, évidemment. J'espère que nous saurons capitaliser sur ces réussites récentes pour stimuler l'innovation et réindustrialiser le pays.

une rente de situation que nous avons dénoncée et qui fait l'objet de critiques régulières dans de nombreuses études économiques ? Je rappelle que les modifications que nous proposons ne font que corriger à la marge certains abus, sans porter atteinte au coeur du dispositif.

puisque l'actuel taux de 30 % sera augmenté à due concurrence des économies réalisées, en supprimant le taux de 5 % au-delà des 100 millions d'euros de dépenses de R&D et en calculant le plafond du CIR au niveau de la holding de tête pour les groupes qui pratiquent l'intégration fiscale.

Quant à l'argument de stabilité fiscale qui a été évoqué, il ne tient pas davantage selon moi. Comme Mme le rapporteur l'a souligné et comme certains collègues l'ont rappelé, le contexte fiscal des entreprises a changé. En outre, le dispositif du CIR n'a pas évolué depuis Le temps d'une évolution est donc venu, d'autant que les études économétriques démontrent qu'une révision même marginale du CIR s'impose pour garantir l'efficacité de la dépense publique. chers collègues, à l'heure où le Parlement est souvent critiqué pour son impuissance, j'espère que nous vous avons convaincus de cosigner et de voter les amendements transpartisans que nous vous proposerons, Vanina Paoli-Gagin et moi-même, au moment de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, afin de renforcer la compétitivité de nos PME et ETI par l'innovation. Au-delà du CIR, je souhaite insister sur une autre mesure qui nous paraît importante pour promouvoir l'innovation dans les PME qui ne font pas encore appel aux dispositifs d'aide à la R&D. À l'instar de ce qui se fait en Belgique, nous proposons d'instituer un « coupon recherche-innovation » de 30 000 euros à destination des PME, dans la limite d'une enveloppe globale de 120 millions d'euros. Ce dispositif permettrait d'élargir le vivier des bénéficiaires des aides à l'innovation à des PME, par la bureaucratie associée au dispositif de soutien à l'innovation. Dans nos circonscriptions, nous avons tous entendu des chefs d'entreprise se plaindre qu'ils n'avaient ni le temps ni les ressources humaines pour remplir les dossiers d'appels à projets. au cours de nos auditions, nous avons constaté que c'étaient souvent les mêmes entreprises qui bénéficiaient des aides publiques d'une année sur l'autre, notamment parce qu'elles pouvaient s'appuyer sur des services juridiques disposant d'une expertise pour remplir ce type de dossiers. Nous avons également été choqués d'entendre que 15 % du montant des appels à projets servirait en réalité à rémunérer des cabinets de conseil chargés de monter les dossiers ! Le « coupon recherche-innovation » vise donc à rétablir une certaine égalité devant les aides publiques en permettant aux PME de se lancer dans un processus d'innovation indispensable pour leur compétitivité future, donc pour leur pérennité,

doit mobiliser la commande publique au service des entreprises industrielles innovantes. Les chefs d'entreprise attendent moins des subventions que des opportunités pour faire croître leur chiffre d'affaires. Or la commande publique représente chaque année 111 milliards d'euros ... Il existe une idée fausse, malheureusement très répandue, selon laquelle les règles communautaires seraient à l'origine de notre incapacité à utiliser la commande publique pour soutenir nos entreprises. En réalité, nous nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues à cause d'une conception rigide et peureuse des règles des marchés publics. D'autre part, le Gouvernement doit renforcer toutes les initiatives de facilitation des démarches administratives et de raccourcissement des délais, afin d'aligner le temps administratif sur le temps économique. En conclusion, si les défis sont grands, je suis, comme Mme le rapporteur, optimiste, car la France dispose des atouts nécessaires pour faire partie des grandes nations innovantes. Le débat d'aujourd'hui a montré une réelle prise de conscience, de la part aussi bien du Parlement que du Gouvernement. Désormais, il nous faut agir collectivement pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques consacrées à l'innovation et, surtout, pour les mettre au service de la réindustrialisation de nos territoires- de tous nos territoires.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire a exacerbé les faiblesses de l'hôpital public, où le manque de lits ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. Nous en avons parlé longuement lors de notre débat mardi : les difficultés éprouvées par le secteur sanitaire, au plus fort de la crise, pour répondre à la demande de soins, témoignent de la défaillance plus large à laquelle fait face, comme dans tant d'autres pays voisins, notre système de santé. La Nation a pu, à cette occasion, témoigner sa reconnaissance au personnel soignant et hospitalier, en première ligne face à la covid-19. Les personnels des établissements médico-sociaux se sont également mobilisés pour maintenir la continuité du lien et des accompagnements, que la situation menaçait de mettre gravement en péril. Ils ont été centraux pour tout notre système de soins- sanitaires et sociaux -si cher à nos valeurs et à notre histoire. La crise sanitaire a suscité dans l'urgence des solidarités nouvelles et a encouragé la mise en oeuvre de prises en charge innovantes. C'est dans les crises que nous sommes le plus créatifs, que les barrières s'abaissent et que les collaborations se lient. Une fois encore, la pandémie nous a démontré la véracité de cette idée.

nous interrogions sur la place que pourraient occuper les acteurs du médico-social dans la nouvelle organisation des soins de demain. Trop souvent, un regard inquiet se porte sur l'hôpital et sur la médecine de ville, comme uniques garants de la continuité des soins. Ceux-ci sont essentiels, c'est certain, et notre groupe saura, dans les mois prochains, défendre avec vigueur leur rôle. Mais ils ne sont pas les seuls ils ne sont pas les seuls pour résoudre le problème grandissant des zones sous-dotées ; ils ne sont pas les uniques relais pour assurer la prévention. Le secteur du médico-social et tous les professionnels qu'il comprend sont au coeur de notre politique du soin dans dans toute sa pluralité et sa complexité. Ses acteurs interviennent dans des domaines variés, tels que celui de l'enfance, du plus grand âge, du handicap, de la protection maternelle et infantile, auprès de personnes en grande difficulté sociale et de santé, ou encore dans le cadre de la protection des majeurs. Il joue un rôle déterminant dans notre société. Un rôle économique, d'abord, en libérant du temps pour les aidants salariés ou en prévenant la désinsertion en prévenant la désinsertion professionnelle des personnels fragilisés par le handicap ou la maladie. Il assume aussi un rôle social de maintien du lien de solidarité, dont la nécessité a été exacerbée durant la crise. Alors que les attentes vis-à-vis de ces personnels sont fortes, et que ceux-ci doivent assurer la prise en charge de la précarité, ils se sentent parfois eux-mêmes précaires. Aussi, comme l'hôpital, le secteur médico-social est-il en proie à des difficultés de recrutement. Je tiens ici à souligner l'effort consenti par le Gouvernement pour un million de professionnels de ces secteurs dont les rémunérations ont été revalorisées, qu'il s'agisse des professions médicales, des professions du soin ou, pour certains secteurs, comme celui du grand âge, des professions de l'accompagnement. accordée dans le cadre du Ségur de la santé, a été élargie également aux professionnels du secteur socio-éducatif dans tous les établissements et services du handicap, de la protection de l'enfance, de l'insertion ou encore de l'hébergement. S'adressant à un public de personnes par définition vulnérables et dépendantes, les acteurs du médico-social occupent une position stratégique dans l'organisation du soin et sont susceptibles d'intervenir à des étapes clés de la prise en charge médicale d'éventuels patients. Face au vieillissement de la population et à l'accroissement du nombre de personnes âgées de plus en plus dépendantes, garantir à celles-ci une prise en charge adaptée à leur état, selon leur degré d'autonomie, permettrait de libérer du temps médical. Il s'agit de favoriser le maintien à domicile des personnes légèrement dépendantes, grâce au renforcement de l'aide à domicile et au financement de l'adaptation des logements.

Garantir une prise en charge adaptée à nos aînés, c'est permettre de mieux vieillir, et c'est encore du temps médical qu'on libère. Je pense aussi à nos enfants, dont les problématiques de santé mentale se font de plus en plus inquiétantes. Les éducateurs spécialisés connaissent les jeunes, ils pourront être des garants d'un diagnostic précoce et ils sont utilement formés à ces enjeux. Je pense encore à nos concitoyens nos concitoyens en situation de handicap, dont l'inclusion dépend aussi de la place donnée aux professionnels du médico-social dans toutes nos structures, qu'il s'agisse d'éducation ou d'emploi. Aussi nous faut-il imaginer de nouvelles formes d'organisation des soins afin d'être, demain, en mesure de proposer, dans les territoires, une offre de soins adaptée aux besoins qui sont exprimés. exprimés. Organiser les soins de demain en collaboration avec les acteurs de nos territoires, c'est donner à chacun toute sa place. C'est laisser la possibilité aux élus locaux de trouver des solutions aux enjeux de terrain qu'ils connaissent si bien. C'est donner aux nouvelles générations de professionnels des possibilités novatrices pour collaborer vers un vivre ensemble inclusif et protecteur. Mes chers collègues, le sujet qui nous occupe aujourd'hui est vaste, mais il existe toujours, dans les questions d'ampleur, des solutions concrètes et, dans les grands débats, de petites victoires.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord remercier le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour de votre assemblée. Je profite de la tenue de ce débat pour saluer les quelque 11 millions de nos concitoyens engagés qui viennent en aide chaque jour aux personnes en perte d'autonomie dans notre pays. Le 6 octobre est, comme vous le savez, la journée nationale des aidants. Ceux-ci ont tout notre respect et méritent une attention constante. Quelle place donner aux acteurs du médico-social dans l'organisation des soins de demain sur nos territoires ? Je veux vous redire le plaisir qui est le mien d'intervenir devant vous sur ce sujet, qui soulève des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre système de santé, tant en matière d'égalité d'accès à la santé sur le territoire que d'attractivité des métiers du médico-social. Avant de parler de demain, ce débat mérite un mot sur hier, avec un constat : la crise sanitaire, qui a été une épreuve collective, a notamment montré combien notre système de soins a besoin de dépasser l'hospitalo-centrisme pour aller vers des coopérations territoriales entre acteurs du soin et du et du médico-social. Le Gouvernement tire toutes les leçons de ce constat. C'est pourquoi le sujet de l'organisation territoriale des soins est au coeur de mon ministère, en lien avec mes collègues François Braun, Jean-Christophe Combe et Geneviève Darrieussecq.

En particulier, le sujet du bien vieillir constituera un axe central de notre action gouvernementale. Il s'agit notamment d'assurer le « virage domiciliaire », en permettant à nos concitoyens de disposer de solutions de maintien à domicile ou de prise en charge dans des structures adaptées à la diversité de leurs situations.

une large concertation avec l'ensemble des acteurs pour faire émerger des solutions concrètes, pragmatiques et adaptées aux besoins des territoires. La crise a agi comme un révélateur de nos faiblesses, mais aussi comme un formidable catalyseur en matière d'innovation technologique et organisationnelle. Partout sur le territoire, des organisations nouvelles ont été déployées, des freins historiques ont été levés et des solutions locales ont été trouvées, en matière d'aller vers, d'accompagnement et de prise en charge. C'est cet état d'esprit que nous souhaitons conserver et promouvoir dans le cadre de ce CNR, pour construire la santé de demain avec l'ensemble des parties prenantes, locales et nationales, dans une logique de confiance, de coopération et de subsidiarité. Pour revenir au coeur même du débat, je voudrais rappeler que le secteur médico-social a d'ores et déjà une place essentielle dans l'organisation actuelle des soins. Je suis convaincue que, dans un avenir proche, la coopération renforcée entre le sanitaire et le médico-social constituera un enjeu clé et pourra apporter et pourra apporter des solutions concrètes aux besoins exprimés par nos concitoyens. Il nous faut donc réinventer la place des acteurs du secteur médico-social dans l'organisation territoriale du soin, au sens du, du, avec des enjeux de sensibilisation, de formation, de coordination, d'accompagnement des professionnels de santé et de prévention, en ce qui concerne notamment Réinventer la place des acteurs du secteur du médico-social dans l'organisation territoriale des soins, c'est aussi, bien entendu, parler de l'avenir des métiers de ce secteur, qui est aujourd'hui le quatrième pourvoyeur d'emplois dans notre pays, et qui s'est fortement mobilisé pendant la crise sanitaire. À ce titre, je tiens une nouvelle fois à saluer l'engagement de l'ensemble des personnels du secteur qui, partout sur le territoire, se sont mobilisés sans relâche pour combattre l'épidémie. Je remercie de même tous ceux qui ont accompagné nos personnes âgées pendant la canicule cet été. Ces métiers essentiels de l'accompagnement et de la prise en charge du médico-social souffrent, comme tous les métiers du soin, de profondes difficultés. Je tiens à rappeler l'importance des efforts financiers réalisés en 2022 en faveur de l'attractivité des métiers de l'autonomie, sous l'effet notamment de l'extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé au personnel des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, avec les accords Laforcade, ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social, qui ont représenté un effort de 3,2 milliards d'euros pour la branche autonomie. Néanmoins, les tensions qui subsistent sur les métiers de l'accompagnement ne se résument pas aux enjeux, légitimes, de rémunération. Il nous faut aller toujours plus loin pour renforcer l'attractivité de ces métiers, améliorer les conditions de travail, accompagner la construction de parcours et de carrières ou encore rénover la formation. C'est aussi l'objet de notre débat ce jour. Aussi l'action du Gouvernement en faveur de l'attractivité des métiers de l'autonomie est-elle guidée par deux grands principes, qui nous permettront de préparer cet avenir. D'abord, simplifier et fluidifier, parce qu'il faut faciliter les démarches à celles et ceux qui veulent s'engager dans ces filières. Puis, reconnaître et valoriser, parce que ces métiers doivent pouvoir susciter des vocations et trouver leur juste place au sein de notre société. Ces principes sont traduits par des mesures concrètes dans le PLFSS. Je pense à l'instauration de deux heures hebdomadaires consacrées au lien social auprès de nos aînés, à la transformation des Ehpad, à la création de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), ou encore aux mesures en faveur de l'amélioration de l'accès à la santé. Mais je voudrais surtout mettre en avant le changement de méthode pour appréhender au mieux les changements de demain. Nous souhaitons poursuivre cet effort, à travers le CNR et l'ensemble de notre action. Dans ce but, j'ai notamment engagé des discussions avec les fédérations représentatives du secteur, dans le cadre d'une réflexion plus globale intégrant les problématiques de formation initiale et continue en santé. Cette méthode, notre méthode, repose sur l'ouverture, le dialogue et la concertation. la concertation. En effet, les réponses doivent être issues des territoires et coconstruites avec l'ensemble des acteurs concernés : les parlementaires que vous êtes, les collectivités locales, les associations, les entreprises,

Quel regard porter sur le vieillissement ? Quelle place donner aux professionnels du médico-social et aux proches ? Quel accompagnement offrir dans nos territoires ultramarins trop souvent sous-dotés ?

à travers le dispositif de validation des acquis de l'expérience. Mais l'organisation des soins de demain nous impose de poursuivre nos efforts. Dans le dernier rapport de l'Insee, il est souligné que, entre 2020 et 2030, le nombre de seniors dépendants âgés de 60 à 74 ans augmenterait de 15 % en Guadeloupe. Au-delà de 75 ans, cette hausse sera de 45 %. Or, actuellement, seuls 5 % d'entre eux vivent en institution, et 6 695 emplois seraient nécessaires en 2030 pour prendre en charge, avec respect et dignité, nos concitoyens âgés. Quelle collaboration mettre en oeuvre demain entre citoyens et professionnels du domaine sanitaire et médico-social pour assurer

déléguée. Monsieur le sénateur, vous rappelez la tradition de solidarité familiale qui est ancrée dans les valeurs et l'organisation de l'accompagnement des personnes dans votre territoire de Guadeloupe.

L'accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap et âgées est un enjeu pour notre société, une ambition pour le Gouvernement, et ce pour l'ensemble du territoire. C'est pourquoi de nouvelles places seront créées dans les services de soins infirmiers à domicile et le modèle de tarification évoluera dans les mois à venir, pour mieux valoriser la prise en soin des personnes les plus dépendantes. C'est aussi pour améliorer le soin à domicile qu'un tarif plancher de 22 euros a été mis en place pour les interventions des services d'aide à domicile qui interviennent dans le cadre de l'allocation personnalisée Vous soulignez aussi le manque d'établissements sur votre territoire pour les personnes qui ne pourraient ou ne souhaiteraient plus vivre à domicile. Un plan d'aide à l'investissement, géré par la Caisse nationale cours : 17 millions d'euros seront ainsi destinés aux territoires d'outre-mer et à la Corse dans le cadre d'un plan de rattrapage visant à la réhabilitation du parc existant, mais également à l'installation de places nouvelles. La parole est

C'est historique et c'est culturel, les fonctions du soin souffrent d'avoir été longtemps, trop longtemps, naturellement exercées par des femmes : moins un métier qu'une occupation, une inclination personnelle, voire une vocation. Ces différentes appréciations rendent invisibles les compétences exercées, la technicité des gestes, la complexité des relations humaines construites avec les personnes vulnérables et leurs familles. La valeur de ce travail est clairement sous-estimée. Si l'on compare les tâches professionnelles de prendre soin à d'autres métiers, qui mettent en jeu une technicité comparable, une aisance relationnelle similaire et l'exercice de responsabilités, l'écart de considération est flagrant, notamment quand on les compare avec des métiers à prédominance masculine. Ce qui découle de cette sous-reconnaissance est évident le cumul de faibles rémunérations et de temps de travail partiels, scindés, le plus souvent subis. Rien ne justifie la persistance d'une telle vision des choses. Madame la ministre, comment le Gouvernement entend-il prendre ses responsabilités

Le secteur médico-social est composé d'une diversité de lieux d'exercice et de métiers, de la petite enfance à la gériatrie, mais toutes et tous vivent la même réalité : le manque de reconnaissance de leur métier.

Or il n'en reste que 309 en France ! Quand on sait les conséquences de la pandémie sur les enfants et les adolescents, il y a de quoi s'inquiéter. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un colloque, que j'organise lundi au Sénat. Madame la ministre, nous sommes face à un abandon institutionnel de ces professionnels et, de fait, de leurs patients, d'autant qu'en excluant nombre de ces professions des revalorisations du Ségur de la santé, le sentiment de dévalorisation de leurs métiers s'est généralisé. Malgré les rattrapages de l'an dernier, les « oubliés » du Ségur existent toujours. Quand allez-vous revaloriser tous ces métiers de la deuxième ligne, madame la ministre ? Enfin, je voudrais attirer votre attention sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur, ainsi qu'à ma collègue Cathy Apourceau-Poly : les aides à domicile. Il y aurait beaucoup à revendiquer, mais je vais centrer mon propos sur le prix de leurs déplacements en voiture qui s'envole depuis la crise en Ukraine et les conséquences sur le prix de l'essence. Allez-vous enfin, madame la ministre, relever le barème kilométrique des aides à domicile de 0,22 euro à 0,35 euro pour permettre à ces personnes de faire face aux difficultés qu'elles rencontrent

Le secteur du grand âge se mobilise face à la transition démographique et la prise en charge médicale et paramédicale des résidents en Ehpad évolue. Ainsi, de nouvelles exigences, utiles et nécessaires, sont venues modifier la pratique des soignants coordination des parcours de soins, concertation, pluridisciplinarité, démarche qualité, etc. Alors que les établissements peinent à recruter des personnels soignants, le marché de l'emploi des secrétaires médicales, des enseignants en activité physique adaptée

Il est donc temps de mettre en cohérence le financement des Ehpad avec les ambitions sociétales, de répondre aux nouveaux besoins des prochaines années et de donner une impulsion au secteur du grand âge de demain. Ainsi, l'intégration de ces professions dans le champ du forfait soins des Ehpad permettrait une application durable et immédiate de mesures favorables aux résidents- contact avec les familles, coordination des soins, etc. -et aux équipes- soulagement des professions en tension ou encore accroissement du temps passé au chevet des résidents.

Toutefois, ce mode de financement n'est pas satisfaisant, puisqu'il ne permet pas d'ancrer ces professionnels dans le fonctionnement de l'établissement de manière durable. Le groupe Union Centriste souhaiterait connaître, madame la ministre, la position du Gouvernement sur l'idée d'intégrer ces professionnels à la section soins des Ehpad de soutenir les personnels médicaux et paramédicaux et de répondre à la pénurie de professionnels, en tenant compte de l'émergence de nouvelles professions au service du soin. La parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice,

Il y a un siècle, seuls quatre Français sur dix atteignaient l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, la France compte 1,5 million de personnes âgées de 85 ans et plus. À l'horizon de 2060, elles seront 5 millions et le nombre de personnes âgées dépendantes pourrait atteindre 2,3 millions. Cette évolution démographique et épidémiologique constitue un défi majeur pour notre société et impose que nous allions plus loin par la mise en place d'un plan ambitieux pour accompagner le vieillissement de la population, domaine dans lequel les professionnels médico-sociaux jouent un rôle essentiel. Or ces métiers souffrent aujourd'hui d'une pénurie croissante et ne parviennent pas à recruter à la hauteur des besoins. Certes, il est indispensable d'améliorer les rémunérations

Actuellement, la gériatrie ne fait pas partie des domaines dans lesquels des infirmiers en pratique avancée peuvent pratiquer. Cette absence de reconnaissance freine le développement de la filière IPA, que ou à domicile, alors qu'il apporterait une véritable valeur ajoutée sur la qualité des prises en charge, l'organisation des soins et la valorisation des professionnels. Cette reconnaissance est d'ailleurs fortement attendue par le secteur du grand âge, comme le rappelle la Société française de gériatrie et de gérontologie. Aussi, madame la ministre, j'aimerais connaître votre position sur la reconnaissance de la spécificité des infirmiers en pratique avancée en gérontologie. La parole est à Mme la ministre

Quand l'accompagnement à domicile par une aide ou une infirmière ne suffit plus, il faut apporter un complément, par exemple un renforcement du temps passé avec la personne, l'intervention d'une diététicienne ou d'une psychologue, la sécurisation du domicile par un ergothérapeute ou encore le renforcement des interventions la nuit.

2019. Les centres de ressources territoriaux qui sont en cours de déploiement présenteront de manière pérenne une offre d'accompagnement renforcé à domicile en alternative à l'Ehpad. objectif est bien de donner corps à la promesse du virage domiciliaire : permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles, même lorsque leur niveau de perte d'autonomie et leurs besoins de soins augmentent. Alors qu'on les orienterait aujourd'hui vers un Ehpad, l'accompagnement renforcé à domicile permettra à ces personnes de rester chez elles plus longtemps.

La demande en personnel est croissante dans ce secteur, de nombreuses offres d'emploi restent vacantes et, chaque jour, des personnes vulnérables ne reçoivent pas les soins nécessaires. Notre société et nos territoires évoluent très rapidement. Les besoins ont changé, la manière d'y répondre également. Il me semble essentiel d'avoir une vision d'ensemble pour répondre aux problématiques du secteur médico-social et repenser l'organisation spatiale des soins de demain. De manière globale, les secteurs médico-social, paramédical et médical doivent travailler main dans la main. Dans ce cadre, la formation, qu'elle qu'elle soit initiale, continue ou de reconversion, est la clé. Et cette formation doit être dispensée au plus près des territoires. J'en veux pour preuve l'implantation à Melun d'une antenne de l'université Paris-Est Créteil. C'est excellent pour notre territoire, surtout lorsque l'on sait que les étudiants s'installent généralement où ils ont étudié. Cela doit être encouragé et développé. De plus, la construction de pôles de santé sur nos territoires est un enjeu et il faut savoir qu'ils sont très souvent associés à des services médico-sociaux. Nous devons donc C'est pourquoi nous devons développer un panel de formations intégrées dans un système complet, équilibré et efficace, qui s'adapte autant aux spécificités de nos territoires qu'aux évolutions démographiques, sans oublier de valoriser ces métiers.

déléguée. Madame la sénatrice, vous avez raison de rappeler l'importance des acteurs du secteur médico-social partout en France- nous ne le dirons jamais assez ! Leur engagement a été particulièrement remarquable lors de la crise du covid-19

ailleurs, il est urgent d'innover, de repenser les outils à la disposition du secteur médico-social de façon différenciée pour chacun des territoires et en corrélation avec le schéma départemental de l'autonomie. Une attention toute particulière doit être portée sur la formation des personnels la mise en oeuvre d'outils de concertation entre l'État, les collectivités locales et tous les acteurs du soin et de l'accompagnement. Il est particulièrement important sur mon territoire, la Guadeloupe, qui est un archipel, coordonner la prise en charge des personnes âgées à travers les dispositifs d'appui à la coordination (DAC) dans le cadre des méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia) en application de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il est également important de rétablir une équité salariale entre les différents personnels du secteur médico-social. provoquent des tensions, mais aussi des difficultés de recrutement dans la plupart des établissements privés à but non lucratif, en particulier pour le secteur associatif, qui prennent en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées

trois secteurs sont en manque de personnel, ce qui aboutit à des politiques publiques essayant de juguler le manque d'attractivité de ces métiers. Pour répondre à ce déficit de vocations, les ajustements sont multiples.

Madame la ministre, avant d'imaginer la place des acteurs du médico-social dans l'organisation des soins de demain, encore faudrait-il sécuriser le périmètre afin que les professionnels des Saad puissent exercer correctement leur métier qui est de prendre soin, en trouvant du sens à leur activité professionnelle. Or le compte n'y est pas. Ainsi, dans le département du Nord, c'est de la survie même des Saad qu'il est question leurs finances sont fragilisées et l'année est pourtant loin d'être terminée. C'est pourquoi nous appelons à des dispositions bordées et soutenables. Sur le plan organisationnel, nous avons déjà voté la fusion

Vous le soulignez à juste titre, la proposition contenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 de dégager deux heures de convivialité pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la nouvelle grille des salaires permettront de mieux reconnaître les métiers et l'expérience

son application en 2023 permettra de mieux valoriser les Ssiad qui prennent en charge des personnes très dépendantes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit aussi une augmentation des places en Ssiad- il faut le souligner. Pour les futurs services d'autonomie à domicile, le forfait coordination déjà en place sera maintenu. Créer les conditions d'un travail en équipe est un levier complémentaire des revalorisations salariales pour la qualité des interventions et la qualité de vie au travail des personnels.

familiale. Les SPTA devront assurer un lien entre les structures, mais leur mise en place se fera en respectant et en s'appuyant, territoire par territoire, sur les organisations qui fonctionnent déjà.

Une grande partie de ces personnes seront en perte d'autonomie et la place des acteurs du médico-social dans l'organisation des soins sera donc de plus en plus importante. Avec le Ségur de la santé, le Gouvernement a prévu d'investir autant dans le secteur médico-social que dans les établissements de santé. Pourtant, les structures qui gèrent les personnes dépendantes, âgées ou porteuses de handicap se trouvent souvent en difficulté, malgré le soutien financier très important des conseils départementaux.

C'est un engrenage, car cela ne permet pas d'assurer l'encadrement suffisant des résidents et entretient des conditions de travail dégradées pour le personnel. Il y a aussi des difficultés face à l'augmentation des charges de de fonctionnement liées à la hausse des prix de l'énergie, des denrées alimentaires, des fournitures, sans oublier les charges de personnel. Ces coûts supplémentaires ont un impact sur la capacité des établissements à investir dans la modernisation du bâti, souvent ancien, des Ehpad publics et contribuent à l'augmentation des tarifs d'hébergement.

avec des places de formation supplémentaires, des dispositifs de formation courte pour les demandeurs d'emploi. Il s'agit également de faciliter l'accès à la formation continue des professionnels en poste, en leur offrant plus de possibilités de bénéficier de la le développement de viviers de recrutement en aidant des employeurs à recruter, notamment avec les vingt plateformes des métiers de l'autonomie, qui facilitent le recrutement et l'intermédiation au niveau départemental. aussi de faire découvrir les métiers du grand âge à de nouveaux publics, notamment les jeunes, en leur proposant des missions de service civique et des stages de troisième, et les demandeurs d'emploi, en travaillant avec Pôle emploi pour leur proposer des formations courtes, des contrats aidés, des périodes de mise en situation professionnelle. les personnes éloignées de l'emploi, les personnes réfugiées, avec des dispositifs pour leur faire découvrir ces métiers. C'est bien en travaillant sur l'image de ceux-ci que nous arriverons à recruter massivement les professionnels dont nous avons besoin.

La revalorisation issue du Ségur de la santé, déclinée ensuite dans le médico-social, a conduit au versement d'une prime par touches successives, après de multiples appels à considérer les « oubliés » du Ségur.

Là où il est censé s'appliquer, la réalité est assez confuse et, malheureusement, il subsiste encore des invisibles du Ségur. Tout l'été, des professionnels ont témoigné de ces injustices, notamment les agents affectés aux missions administratives ou logistiques dans les établissements. Cette segmentation est injuste et délétère. Injuste, car les personnels savent que, sur le terrain, ce cloisonnement n'a pas lieu d'être : un agent d'accueil en Ehpad est au contact des résidents et de leur famille ; un agent de ménage travaillant dans un établissement de l'aide sociale à l'enfance (ASE) participe à la mission éducative quand il s'assure du respect des règles de propreté. Délétère aussi, car elle indique la porte de sortie à des personnels formés et compétents, rapidement employables dans le privé. Certes, ces tensions ne dépendent pas que de l'État, certaines collectivités tardant aussi à financer leur part de cette revalorisation, mais il est de votre devoir, madame la ministre, d'orchestrer l'entrée en application Ma question est simple : le Ségur pour toutes et tous, c'est pour quand ?

Les pouvoirs publics incitent depuis plusieurs années à la mise en place d'une médecine de « parcours »- de santé, de soins, de vie -, à même de renforcer la prise en charge des patients et des résidents sur tout le territoire et de décloisonner les secteurs. L'objectif affiché est de prévenir, de soigner et d'accompagner de manière globale et continue les patients et les résidents, au plus près de chez eux. Cet objectif suppose une bonne répartition des structures sanitaires, médico-sociales et ambulatoires sur le territoire national, mais aussi la complémentarité efficace des professionnels de ces structures. Cet objectif doit aussi accompagner un virage domiciliaire, qui répond aux souhaits d'une part grandissante de la population. Dans ce contexte, les acteurs du médico-social ont donc un rôle à jouer dans l'organisation de l'offre de soins, et notamment dans l'offre de soins de demain, qui va devoir prendre en compte le vieillissement de la population. Compte tenu des difficultés de recrutement du secteur médico-social aujourd'hui, des médecins aux aides-soignants, cette participation à l'organisation des soins de demain suppose néanmoins de faire bouger les lignes pour renforcer l'attractivité du secteur. Ma question, madame la ministre, portera sur l'architecture budgétaire, et donc, indirectement, sur les moyens. Les dépenses relatives aux soins à domicile, à savoir celles du virage domiciliaire, relèvent de deux enveloppes différentes, répondant à des logiques de régulation différentes différentes : dotation limitative pour les services de soins à domicile ; enveloppe ouverte pour les actes infirmiers, pour me limiter à ces exemples. Comment faire, alors, pour que cette architecture institutionnelle ne soit pas un frein à la participation du médico-social à l'organisation des soins de demain

des aides à domicile. On voit bien que l'articulation entre les services à domicile et les actes infirmiers, deux domaines différents et complémentaires, est nécessaire. À nous d'inventer les modèles de financement qui permettent une prise en charge globale à domicile.

Les acteurs du médico-social sont divers et variés. En plus des acteurs éducatifs, nous y retrouvons des soignants- aides-soignants, infirmiers, médecins généralistes, psychiatres -, et des paramédicaux- orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues. Les dirigeants de ces structures ont depuis longtemps compris l'intérêt du maillage territorial et de la coordination du parcours des personnes accompagnées par leurs structures : parcours éducatif, parcours de soins, maillage et partenariat. Les communautés professionnelles territoriales de santé et médico-sociales pourraient être l'une des réponses. Il s'agirait de s'appuyer sur ce secteur pour renforcer les soins de demain sur nos territoires,

En revanche, dans un contexte de traitement inégalitaire entre le sanitaire et le médico-social au regard des revalorisations Ségur et Laforcade, comment comptons-nous donner envie à ce secteur de s'engager dans un nouveau défi portant sur le soin ?

qui se sont entendus pour le créer. Je suis intimement convaincue que ce dispositif ne peut fonctionner que s'il est créé par les professionnels, pour les professionnels, au seul bénéfice de l'accompagnement de nos concitoyens.

doit également permettre d'accroître l'efficience du soutien à l'autonomie. Elle est aussi la promesse d'une solidarité renforcée pour l'ensemble des citoyens nécessitant

À la suite de la création, en 2007, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, il n'y a pas été créé de maison territoriale des personnes handicapées, analogue des maisons

personnes dont les compétences permettent d'assurer pleinement les missions d'une MDPH au sein de la direction de l'autonomie. Cette direction est organisée de manière à assurer sa mission auprès des personnes en situation de handicap, mais aussi en perte d'autonomie. À l'instar de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, mon territoire doit pouvoir rapidement migrer vers le dispositif de MTA. Cela nécessite une modification du code de l'action sociale et des familles,

déléguée. Madame la sénatrice, l'équité dans l'accès aux droits pour toutes les personnes âgées et en situation de handicap est une nécessité défendue fermement par le Gouvernement. Cette équité demande de pouvoir décliner les organisations des maisons départementales des personnes handicapées et les services du département en fonction du territoire. on ne propose pas un accueil de proximité de la même façon dans les Hauts-de-Seine, en Haute-Loire, en Guyane, ou à Saint-Martin. La mise en place, dès 2006, d'une maison territoriale de l'autonomie à Saint-Pierre-et-Miquelon résulte résulte d'un choix fort de cette collectivité. D'autres travaux sont conduits par les collectivités d'outre-mer, comme il est prévu dans la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique Dès maintenant, pour garantir l'équité de traitement pour les personnes, les professionnels du pôle autonomie de Saint-Martin peuvent s'appuyer sur les outils mis à leur disposition par la CNSA : guides, webinaires d'information et échanges de bonnes pratiques. On peut saluer le suivi individualisé et personnalisé proposé aux habitants âgés ou en situation de handicap de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon par les équipes des collectivités, qu'il s'agisse d'une maison territoriale de l'autonomie ou d'un pôle social.

Un tiers de la population française vit désormais dans un désert médical ; dans le Loiret comme dans plus des trois quarts de nos départements, la densité médicale a diminué en 2021. Sans surprise, la pyramide des âges des praticiens assombrit un peu plus encore ce paysage.

Le modèle de cette profession mérite notre attention : il peut nous inspirer si l'on veut atténuer les difficultés que rencontrent des acteurs du secteur médico-social. Contraints de composer avec des moyens limités, des revenus souvent modestes et un système de formation inadapté, la majorité des professionnels du secteur regrettent de n'être ni considérés ni reconnus. Dès lors, madame la ministre, votre éclairage est espéré sur plusieurs points. En attendant de retrouver un nombre de professionnels de santé en cohérence avec les besoins de nos concitoyens, prévoyez-vous d'étendre la délégation de certaines compétences aux professionnels du médico-social ? Si oui, pouvez-vous préciser les actes concernés ?

vous m'interrogez sur l'attractivité des métiers dans le secteur médico-social ; vous avez commencé par rappeler le nombre de médecins que nous avons perdus en quelques années. C'est bien parce que nous avons perdu 10 000 médecins que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.

Les métiers du lien social souffrent aussi de leur faible attractivité. Afin d'y répondre, je le redis, nous avons déjà mené un nombre important d'actions. Nous avons engagé un effort de 4 milliards d'euros en année pleine pour l'ensemble des professionnels du secteur social et médico-social. On compte

M. Hugues Saury, pour la réplique. Madame la ministre, ce que l'on constate aujourd'hui, ce sont de grandes difficultés à recruter, de nombreux arrêts de travail, des démissions et des demandes de rupture conventionnelle, un sentiment de lassitude et de frustration, enfin une affirmation exacerbée des revendications d'ordre socio-économique autour de la vie chère et du bas bas niveau de pouvoir d'achat. Je doute que votre réponse appelant à changer de regard ne parvienne à rassurer les acteurs du médico-social ! Pendant ce temps, l'hémorragie continue. Or, ne nous y trompons pas, l'avenir de notre système de soins dépend aussi de notre capacité à rendre attractifs ces métiers essentiels dont l'utilité sociale est reconnue. En conclusion du

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, en guise de conclusion, saluer la tenue de ce débat au sein de notre assemblée. Les propositions concrètes qui en ressortent témoignent de l'intérêt que nous, législateurs,

de l'égal accès, sur tous nos territoires, à ces soins de demain sont autant d'enjeux que de solutions possibles. Nous sommes au coeur de la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées,

Leur rôle est au coeur de la République, comme la crise sanitaire l'a encore une fois démontré. Aux côtés des soignants, ils ont été aux avant-postes, mobilisés 24 heures sur 24 pour maintenir la continuité du lien, offrir un accompagnement digne à nos concitoyens les plus vulnérables et gérer, bien souvent, des situations d'urgence. Cela a été dit, ces femmes et ces hommes sont indispensables, parce qu'ils contribuent au maintien des liens de solidarité et au développement de la vie sociale du pays. Ils sont présents dans tous les territoires et dans tous les domaines de l'intervention sociale ceux du grand âge et de la politique du handicap, celui des personnes rencontrant des difficultés sociales et, bien sûr, celui de la protection de l'enfance.

Ces métiers, que nous pourrions qualifier de vocations- éducateurs spécialisés, assistants maternels, aides-soignants, éducateurs de jeunes enfants -, sont au coeur de notre modèle social, puisqu'ils ont un impact sur la vie et sur l'avenir de celles et de ceux qu'ils assistent. Le constat est clair et unanimement partagé, que l'on traite de la protection de l'enfance, du grand âge ou de la politique du handicap : le secteur médico-social souffre. Il souffre d'un manque d'attractivité- vous l'avez rappelé, madame la ministre -, d'un manque de reconnaissance et, par conséquent, d'une pénurie alarmante. Celle-ci a bien sûr des conséquences directes sur les travailleurs sociaux, puisque leur mission est entravée, mais aussi sur les publics fragiles. Concrètement, je pense aux enfants placés sous protection qui n'ont même plus la possibilité de se rendre en visite médiatisée avec leurs parents, faute de professionnels pour les accompagner.

Je pense à l'épuisement des travailleurs sociaux dans certains foyers de l'enfance, qui ont pour mission de gérer, parfois seuls, 40 enfants placés sous protection et devant donc faire l'objet d'une attention toute particulière. Nous, parents ou grands-parents, serions incapables de mener efficacement cette mission. Dès lors, comment un travailleur social, aussi dévoué soit-il, pourrait-il assumer correctement la mission que nous lui confions ? À cet égard, je souhaite saluer l'action du Gouvernement qui, conscient de ces difficultés, décrétera un taux et des normes d'encadrement qui permettront de soulager les travailleurs sociaux et, par ricochet, de mieux protéger les enfants. Mes chers collègues, dans tous les centres de loisirs des 36 000 communes de notre pays, un taux d'encadrement est fixé, qui protège les enfants et sécurise le personnel périscolaire. Il apparaît donc urgent d'établir des règles similaires dans les foyers de l'enfance, alors que nous savons qu'un enfant sur quatre pris en charge par l'aide sociale à l'enfance est en situation de handicap. La revalorisation historique des métiers du secteur médico-social, dont le Gouvernement a pris la décision en février dernier et que nous avons tous soutenue, témoigne de la reconnaissance par l'État du rôle essentiel des travailleurs sociaux dans le soin et l'accompagnement de nos concitoyens les plus vulnérables. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui prévoit près de 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le secteur médico-social, apporte également des solutions concrètes. Je pense notamment à l'effort important en faveur de l'attractivité des métiers de l'autonomie afin de renforcer la qualité et l'offre d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. d'assurance maladie (Ondam), qui continuera sa forte progression en 2023 : une hausse de 3,7 % hors dépenses liées à la crise sanitaire. Les mesures prévues dans ce PLFSS traduisent notre volonté partagée de bâtir une société plus inclusive pour nos concitoyens en situation de handicap, par la poursuite de l'investissement en faveur de la scolarisation des enfants en situation de handicap et les mesures spécifiques concernant l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Nous le remarquons sur tous nos territoires, les professionnels du secteur médico-social ont toute leur part dans l'organisation des soins de demain, parce que le soin inclut non seulement le sanitaire, mais également le social, parce qu'accompagner est aussi une manière de soigner. Pour conclure, je souhaite une nouvelle fois saluer la tenue de ce débat et remercier Mme la ministre et l'ensemble des orateurs des groupes pour la qualité de nos échanges. Ces enjeux, nous le savons, sont d'une importance cruciale. Ils ont trait à notre modèle social, à l'égalité des chances, à notre conception de la solidarité nationale. Nous devrons les traiter ensemble durant les mois et les années à venir et le Sénat, chambre des territoires, devra y prendre toute sa place aux côtés du Gouvernement, des acteurs locaux et du monde associatif.